et ce, bien qu'il soit présent dans le lexique de la loi française depuis 1995. Ce principe a constitué une plus-value admirable au service de la protection de l'environnement dans l'action publique. La précaution vise la prévention des risques, quand les connaissances techniques et scientifiques sont insuffisamment précises. Mais c'est ce principe qui a conduit à interdire l'utilisation d'un certain nombre de produits qui ne disposaient d'aucune alternative viable, parfois en l'absence de certitude scientifique sur leur dangerosité.

Or nous avons justement besoin d'innovations scientifiques pour agir contre le changement climatique et au profit de la viabilité de notre modèle économique et industriel. La question sanitaire étant fréquemment instrumentalisée pour interdire certaines pratiques, il est ici proposé de transformer, dans la Charte de l'environnement, le principe de « précaution » en un principe de « prudence responsable ». En effet, lorsqu'il neige, la précaution est de ne pas rouler, alors que la prudence préconise de rouler, mais moins vite qu'à l'accoutumée. Sur le fondement de ce nouveau principe, aucune pratique ne saurait être interdite, lorsqu'elle contribue à la richesse nationale, si elle ne dispose pas d'une solution de substitution et s'il n'existe pas une probabilité scientifiquement étayée de dangerosité.

Ce principe serait défini par l'obligation, pour les autorités publiques, de mettre en oeuvre des procédures d'évaluation des risques et d'adopter des mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation d'un dommage affectant de manière grave et irréversible l'environnement, non plus lorsque la réalisation d'un dommage est possible, quoique « incertaine en l'état des connaissances scientifiques », mais lorsque sa « probabilité de survenue » est « scientifiquement étayée En réalité, on peut considérer que cet amendement est satisfait par le droit en vigueur, car le principe de précaution n'impose pas de parer à la réalisation de dommages imaginaires ou purement spéculatifs : il faut que la possibilité d'un dommage existe, autrement dit que ce dommage ait un certain degré de probabilité, étayée par des faits. Tout dépend naturellement du degré de probabilité exigé. En 2005, le Constituant a posé un principe équilibré : s'il existe une probabilité de dommage, même légère, les autorités publiques doivent, d'une part, se mettre en mesure d'évaluer plus précisément cette probabilité, d'autre part, prendre des mesures provisoires et proportionnées. La commission ne souhaite pas toucher à cet équilibre. Retrait ou avis

démontre, à l'évidence, qu'il n'y a pas toujours d'accord sur les mots ... Nous estimons qu'il constitue une régression par rapport à la Charte

au juge constitutionnel, alors qu'il conviendrait à notre sens de renforcer l'assise des principes de l'environnement dans le bloc de constitutionnalité. En effet, la fragilité de certaines décisions du Conseil constitutionnel tient notamment à ce que certains principes généraux du droit de l'environnement formulés à l'article L. 110-1 du code de l'environnement ne disposent pas d'une valeur constitutionnelle, mais d'une simple valeur législative et que ces principes mis en balance avec d'autres principes constitutionnels comme la liberté d'entreprendre sont appelés à s'effacer.

de la Charte de l'environnement pourraient fournir des points d'appui pour faire évoluer la jurisprudence du Conseil constitutionnel et par conséquent améliorer concrètement la préservation de l'environnement et la prise en compte des enjeux climatiques, en envoyant un signal clair, non seulement à nos concitoyens, notamment à ceux qui ont participé à la Convention citoyenne, mais également À défaut, la réforme qui est ici proposée, amendée ou non par le Sénat, ne serait que gesticulation et manipulation démagogique, sans aucune utilité concrète ou directe.

il a considéré que le législateur « ne saurait priver de garanties légales le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé consacré par l'article 1 de la Charte de l'environnement », que « les limitations portées par le législateur à l'exercice de ce droit ne sauraient être que liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par un motif d'intérêt général et proportionnées à l'objectif poursuivi

largement, en matière de droits fondamentaux. Les pouvoirs publics doivent être en mesure de prendre les dispositions rendues nécessaires par l'intérêt général ou par d'autres exigences constitutionnelles, même si cela implique dans certains cas de revenir sur des dispositions prises pour la protection de l'environnement.

sur l'article. Depuis le début de la pandémie de covid-19, chaque pays compte ses victimes par milliers. En France, depuis mars 2020, on dénombre plus de 106 000 morts. Depuis plusieurs semaines, l'Inde et le Brésil entassent, chaque jour, les corps par milliers. Notre seule arme pour accéder à l'immunité collective, c'est le vaccin. Ce vaccin est un bien commun mondial, un bien commun qui ne peut être la propriété de personne, dès lors que nous en avons tous besoin pour vivre. À ce titre, nous devons favoriser son accès pour tous. tous. Est-il acceptable de laisser les logiques économiques l'emporter sur la santé humaine ? Nous pensons que non. Joe Biden et l'Union européenne ont répondu au cri d'alarme de l'Inde et de l'Afrique du Sud, en se prononçant en faveur de la levée des brevets sur les vaccins. Ces vaccins ont été très largement financés par les contribuables, puisque près de 7 milliards de dollars ont été distribués aux laboratoires par les États-Unis et l'Union européenne pour financer la recherche. À cela s'ajoutent plusieurs centaines de millions de doses de vaccins achetées par les pays. Et c'est aussi grâce à des dizaines d'années de recherche publique, bien commun de la connaissance, que ces vaccins ont pu être découverts. On peut donc considérer que les vaccins sont des biens communs financés très largement par des puissances publiques dans l'intérêt de l'humanité. Il est nécessaire que la France se positionne pour faire de ces vaccins des biens communs mondiaux. Notre espoir de retour à la vie normale réside dans la vaccination pour tous. D'après les chercheurs, cette pandémie ne sera pas la dernière que l'humanité devra affronter. Les futurs vaccins et traitements devront aussi être considérés et gérés comme des biens communs

la France ne garantirait plus la préservation de l'environnement, mais préserverait simplement l'environnement et la diversité biologique. Elle ne lutterait plus contre le dérèglement climatique, mais agirait simplement contre celui-ci. Au-delà des formules retenues et de l'implication juridique concrète de ces modifications, nous faisons un constat simple : le Sénat a joué le rôle que l'on attendait de lui en éloignant l'idée même de toute réforme constitutionnelle, condamnant ce projet de loi constitutionnelle à la navette permanente, sauf à recourir à l'alinéa 3 de l'article 89, c'est-à-dire à passer par le Parlement réuni en Congrès pour opérer cette modification de la Constitution, une voie qui nous semble largement préférable. Le Sénat aura ainsi fait le choix d'être le meilleur alibi du Président de la République pour un nouveau renoncement qui laissera un goût amer,

favoriser » apparaît peu ambitieux. En effet, comme l'a rappelé le Conseil constitutionnel dans une décision du 24 avril 2015, l'alinéa de l'article 1 qui dispose que la loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux ne crée pas un droit ou une liberté garanti au sens de l'article 61-1 de la Constitution. Mes chers collègues, vous nous amusez avec ces guerres sémantiques, qui masquent mal la régression des politiques publiques environnementales. Le Sénat est toujours d'accord avec la majorité présidentielle quand il s'agit de réduire le droit de l'environnement.

Charles, réveille-toi ! Nous sommes devenus fous ! » Telle est l'injonction que nous pourrions adresser au fondateur de la V République. La défense de l'environnement est quelque chose d'important, et même d'essentiel. Chacune et chacun, ici, en est convaincu. Pour la plupart d'entre nous, dans nos fonctions d'élu local, quand nous en avons, nous essayons de mettre ces questions au coeur de notre action. Pour autant, faut-il toucher à la loi fondamentale ? Faut-il changer notre Constitution en fonction de ces enjeux ?

travers les travaux de la Convention citoyenne pour le climat, je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit par différents orateurs, mais je m'interroge à mon tour : les commissions « environnement » de l'Assemblée nationale et du Sénat ont-elles moins de légitimité que des citoyens tirés au sort pour réfléchir sur ces grands enjeux ?

Monsieur le rapporteur,

préserve l'environnement ainsi que la diversité biologique et agit contre le dérèglement climatique dans des conditions prévues par la Charte de l'environnement de 2004. L'intérêt de la rédaction, au-delà des analyses qui ont été faites depuis tout à l'heure sur la proposition gouvernementale, c'est d'établir à nouveau une articulation claire

à rappeler le rôle central de la Charte de l'environnement à l'article 1de la Constitution, je le vois comme une incitation à mener des politiques publiques plus ambitieuses dans le cadre sécurisant de la dynamique conciliatrice du développement durable- préservation de l'environnement, développement économique et progrès social -, sans pour autant créer de hiérarchie entre les principes constitutionnels ni d'incertitude quant à leur responsabilité. Enfin, il y a un aspect symbolique en faveur de la préservation de l'environnement, de la diversité biologique et contre le dérèglement climatique. C'est un sujet qui est cher à la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable,

Monsieur le garde des sceaux, on ne perd jamais son temps, le dimanche matin, à lire le journal. On en a généralement pour son argent Avant même que le Sénat n'examine ce texte en séance publique, ici dans l'hémicycle, avant même, d'ailleurs, que

la révision et le référendum. C'était l'accusation lancée par un certain nombre de porte-parole, j'imagine, de l'exécutif et du Président de la République.

et il a également été suggéré par le Conseil d'État. Si nous le retenons, c'est pour deux raisons que je tiens à rappeler. D'abord, le verbe « garantir », c'est l'introduction du virus de la décroissance dans notre Constitution

Ce principe permettrait de consacrer une obligation positive pesant sur l'État quant aux exigences de protection de l'environnement qu'il s'est lui-même fixées. L'objectif d'amélioration constante de l'environnement n'a aujourd'hui qu'une valeur législative, inscrite au 9° du II l'article L. 110-1 du code de l'environnement Le principe de non-régression, selon lequel la protection de l'environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement, ne peut faire l'objet que d'une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment Afin de renforcer sa portée juridique et d'élargir son champ d'application, ce principe doit être élevé au rang constitutionnel, dans le but de lui conférer une valeur égale à celle des principes constitutionnels de droit de propriété et de liberté des entreprises, généralement utilisés pour autoriser la mise sur le marché, par exemple, des néonicotinoïdes et de certains produits phytosanitaires extrêmement nocifs pour la santé et l'environnement. La France pourrait ainsi être juridiquement mieux armée pour se conformer aux objectifs instaurés par l'accord de Paris et, plus généralement, à ses engagements internationaux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de promotion de la résilience.

Mettons une petite couche de vernis vert sur le bilan et les Français n'y verront que du feu : voilà à quoi ressemble ce projet de loi constitutionnelle. C'est confondre la Constitution avec un tract de campagne Mais les Français n'ont pas la mémoire courte ! Ce gouvernement, c'est celui qui garantit l'utilisation, même provisoire, je vous le concède, des néonicotinoïdes et du glyphosate, l'artificialisation et le forage des sols, la persistance du chlordécone, la multiplication d'accords bilatéraux de libre-échange sans clause environnementale. C'est celui qui a affaibli les propositions de la Convention citoyenne pour le climat, quand il ne les a pas tout simplement effacées. Eh oui ! Mes chers collègues, voilà que ce même gouvernement s'estime, cette fois-ci sans filtre, lié à la lettre même d'une proposition de cette convention, une proposition que nous partageons, à savoir élever la protection de l'environnement au rang de garantie constitutionnelle. Ce débat constitue aussi une occasion rare pour le Parlement d'enrichir notre arsenal constitutionnel en matière de protection de l'environnement. Cela fait plus de 15 ans que le peuple français n'a pas été consulté. Cependant, la démocratie impose que ce référendum ne se réduise pas à un symbole dans une logique purement plébiscitaire. On aurait pu espérer l'inscription de la règle verte, du principe de la non-régression ou encore l'introduction d'un véritable crime d'écocide, mais le Gouvernement n'affiche aucune volonté de débat ouvert, de travail collectif. seulement faire endosser au Sénat- je crois que tout le monde l'a bien compris -, la responsabilité de l'échec d'une réforme constitutionnelle. Cette dernière année de mandat porte décidément la marque des manigances et des faux-semblants. La ficelle est un peu grosse Oui ! Non ! Oui, mais non ! Voilà à quoi ressemble la politique du Gouvernement, notamment pour la levée des brevets sur les vaccins. Non ! Oui ! Peut-être ! On ne sait pas ! C'est la même chose pour cette réforme de la Constitution. Pas de référendum, référendum, puis nouveau renoncement Monsieur le garde des sceaux, votre valse à trois temps se joue au détriment de nos compatriotes, et si vous aviez voulu plomber cette réforme constitutionnelle, vous n'auriez pas fait mieux. En tout cas, l'absence d'un vote en termes identiques lors de cette première lecture ne fait pas obstacle à la tenue du référendum.

Je conclus : l'ensemble des biens communs mondiaux, au rang desquels figurent notamment le climat, l'eau, la santé, doivent être reconnus dans la Constitution. La France en sortirait grandie, monsieur le garde des sceaux, dans le prolongement du rôle qu'elle a joué dans les négociations sur la COP21 en décembre 2015 pour faire aboutir le premier accord universel sur le changement climatique.

de l'environnement. » Nous savons tous que la Charte de l'environnement a valeur constitutionnelle, puisqu'elle fait partie du bloc constitutionnel. Dans l'absolu, votre amendement me semble satisfait, indépendamment du fait que vous conserviez le verbe « garantir Enfin, sur l'amendement n° 11, c'est également un avis défavorable. Je rappelle que la notion « d'ensemble des biens communs mondiaux » reste encore trop floue pour être inscrite

juristes. M. Bas disait que personne n'avait le monopole de l'écologie. C'est vrai, mais personne non plus n'a le monopole de la perfection juridique ! D'ailleurs, Mme la sénatrice Boyer a souhaité d'autres mots que ceux que la commission a retenus. Cela fait partie du débat démocratique.

objet de remplacer l'article en débat par un autre projet, en réalité, avec l'emploi de la formule « préserve l'environnement ». Je ne peux qu'être défavorable à ce projet s'il tend, comme je le crains, à vider de sa substance l'avancée proposée par la Convention citoyenne

la rendant purement symbolique. En effet, cela n'ajouterait rien à ce que prévoit déjà la Charte de l'environnement, hormis la notion de dérèglement climatique, que nous proposons nous-mêmes. Vous considérez que l'intérêt de votre rédaction est d'opérer un renvoi à la Charte de l'environnement, mais un tel renvoi existe déjà dans le préambule de notre Constitution. s'ils étaient adoptés, fragiliseraient le droit applicable en matière environnementale en affirmant que la France préserve l'environnement « dans les conditions prévues par la Charte de l'environnement Vous semblez exclure toute autre norme, et en particulier le code de l'environnement : or les règles applicables en matière de protection de l'environnement ne sont pas toutes prévues dans la Charte. À l'inverse, le projet du Gouvernement apporte une véritable plus-value au droit actuel grâce à l'emploi du verbe « garantir »,

une quasi-obligation de résultat à assurer la préservation de l'environnement, ou, si vous préférez, une obligation de moyens renforcée. L'intensité de l'engagement ainsi créé pourrait être la source d'un élargissement de la responsabilité pour faute de l'État, mais c'est à ce prix que le renforcement de l'action des pouvoirs publics se concrétisera. C'est une exigence impérieuse au regard de la dégradation actuelle de la situation, que vous soulignez vous-mêmes. Pour ces raisons, le Gouvernement ne peut être, en l'état, que défavorable à ces amendements. Puisque j'ai introduit mon propos en rassurant tout le monde

J'avais lu notamment que ce n'était pas la peine de venir ici. Je suis quand même venu, parce que je crois dans la démocratie, et je crois, je l'ai d'ailleurs déjà démontré, que l'on peut se rejoindre sur un certain nombre de textes, au-delà de ce qui peut nous séparer, grâce à un véritable travail constructif.

qui veut intégrer le principe d'amélioration constante, aussi appelé principe de non-régression. Je me suis expliqué longuement déjà sur cette question. Enfin, avec l'amendement n° 11, M. Kanner souhaite intégrer dans la Constitution la notion de « biens communs mondiaux

monsieur le président, pour indiquer à la Haute Assemblée que nous avons parfaitement connaissance du code de l'environnement, mais qu'il y a aussi un principe de hiérarchisation des normes.

les travaux qui ont été réalisés par 150 citoyens. C'est une procédure de jury citoyen qui est utilisée dans beaucoup de démocraties et qui vient compléter la démocratie représentative. À ce titre, il faut la prendre au sérieux.

Ce que laisse entendre le Gouvernement, ou ce qu'il laisse suggérer, ou ce que l'on pourrait comprendre, c'est que, alors que la navette pourrait se poursuivre, elle serait arrêtée ou elle pourrait être arrêtée par le Président de la République, qui ferait endosser la responsabilité de cet échec au Sénat. C'est cette posture qui n'est pas tolérable Sur la question du gouvernement des juges, j'entends les craintes, mais je suis assez kelsénien et je sais une chose : c'est que nous avons tous été contents que, d'une certaine façon, le juge constitutionnel prenne toute sa place en France.

explication de vote. Comme nous l'avons vu, le Sénat a vidé ce texte de sa substance. Il n'est pourtant pas nécessaire de rappeler la réalité du réchauffement climatique et de la dégradation de l'environnement. La situation est plus que préoccupante, menaçante, et les responsables politiques que nous sommes ont une seule mission : trouver des solutions et les mettre en oeuvre. Cette inscription constitutionnelle aurait permis clairement l'engagement écologique du Gouvernement et du législateur. En cette période électorale, la majorité sénatoriale n'avait nulle envie de faire un cadeau au Gouvernement ; pourtant, ni les profits, ni les dividendes, ni la prospérité économique ne seront en mesure d'arrêter la destruction de la planète ! Les jeunes, eux, ont compris l'urgence. C'est pour cette raison qu'ils sont des dizaines de milliers à descendre dans la rue pour réclamer des garanties et une lutte véritable contre le dérèglement climatique. Dans la version retenue par le Sénat,

trahi la demande de la Convention citoyenne pour le climat, qui, selon la majorité sénatoriale, était une manière de faire primer l'écologie aux dépens de l'économie. Ce projet de loi Le texte adopté par le Sénat sera différent de celui de l'Assemblée nationale. C'est quasiment acté : il n'y aura pas de référendum. Le Président Macron a sûrement d'autres préoccupations en cette période riche en scrutins ... La faute à qui ? À tous ceux qui ne voulaient pas que ce projet aboutisse. Une fois de plus, l'écologie a été sacrifiée. À certains, elle ne sert, de temps à autre, qu'à verdir un peu les bulletins de vote !

face à une terrible crise écologique, qui tue des centaines de milliers de personnes chaque année à travers le monde. On sait que la dégradation de l'environnement est devenue l'une des grandes atteintes aux droits de l'homme.

sans filtre. Nous ne voterons donc pas cette version édulcorée par la droite, qui, de son aveu même, ne souhaite pas de nouveaux effets juridiques et qui renonce à toute ambition climatique pour notre Constitution. Chers collègues de la majorité sénatoriale, vous évoquez souvent le risque d'incertitude et d'instabilité juridiques qu'induit la rédaction initiale.

Vous aviez l'occasion d'en appeler au peuple pour engager, enfin, un grand débat démocratique au sujet de l'avenir climatique de notre République. Vous aviez l'occasion de faire trancher par les Françaises et les Français ce vrai choix de société : pour ou contre un avenir durable garanti par notre Constitution. Vous avez préféré le renoncement. Vous reculez face au défi démocratique.

devront d'agir positivement pour préserver l'environnement et la biodiversité et pour lutter contre le changement climatique. Ce n'est pas rien. Effectivement, c'est contraignant. Mais c'est une avancée majeure, à laquelle on ne peut décemment pas s'opposer, surtout quand on clame haut et fort que l'écologie n'appartient pas à un parti et que tout le monde souhaite protéger l'environnement. Dès lors, cessez de proclamer et agissez, en votant ce texte en l'état. Sinon, cela signifie que vous ne souhaitez pas voir la République agir positivement, en toute circonstance, pour l'environnement. Cela signifie que vous avez d'autres priorités et que vous préférez défendre une somme d'intérêts privés plutôt que l'intérêt général, scientifiquement admis par les chercheurs du monde entier. Dans ce cas, il faut tout simplement l'assumer. Cette obligation d'action est une première étape, mais elle ne saurait suffire. Agir pour préserver un environnement déjà partiellement dégradé, c'est stopper l'hémorragie. Toutefois- j'y insiste -, il faut aller beaucoup plus loin et agir pour améliorer constamment l'environnement. C'est une traduction constitutionnelle du principe de non-régression du droit environnemental.

selon votre analyse, le terme « garantit » « faciliterait l'engagement de la responsabilité des personnes publiques », voire « attribuerait une forme de priorité à la préservation de l'environnement ».

Mais votre souhait de modification montre bien qu'au contraire vous l'analysez comme une mesure forte, ayant un impact réel, que vous cherchez à atténuer. Le terme « garantit » vous fait peur, autant que l'idée de soumettre au référendum une modification issue de la démocratie participative.

Mais ce que vous nous proposez, c'est d'écrire, dans la Constitution, que la France préserve l'environnement dans les conditions prévues par la Charte de l'environnement.

Le scrutin est clos.

a été présenté en mai 2019 par nos collègues Ronan Dantec et Jean-Yves Roux. Sa conclusion est sans appel : la France doit « se préparer à absorber un choc climatique inévitable Ce dérèglement sera lourd de conséquences : aggravation des risques naturels, surmortalité liée aux vagues de chaleur ou à la pollution, propagation des maladies, stress hydrique, dangers pour l'agriculture et l'alimentation, Adopté à l'unanimité, ce rapport formule des propositions visant à amplifier l'effort d'adaptation de la France face aux défis sanitaires, économiques et écologiques que pose le changement climatique, par l'accompagnement des territoires, l'adaptation du bâti et de l'urbanisme, la réduction des tensions portant sur les ressources hydriques ou encore l'adaptation de notre modèle agricole. Aussi, cet amendement vise à préciser dans la Constitution que, pour lutter contre le dérèglement climatique, il faut également combattre ses conséquences, qui menacent la vie quotidienne de nos concitoyens.

Ce concept a été proposé par une équipe internationale de vingt-six chercheurs, dans le cadre de travaux publiés en 2009, et est d'ores et déjà utilisé par de grands groupes industriels privés, qui cherchent à confronter leur impact sur l'environnement à la capacité de notre planète à l'absorber. L'objectif de l'inscription de ce concept dans la Constitution est clair : notre société ne doit pas évoluer au détriment des capacités de notre planète, de ses ressources naturelles et de leur capacité éventuelle de renouvellement.

Ainsi, cette inscription dans la Constitution solidifierait toute démarche d'inscription dans le droit de limites chiffrées d'émission de CO2, de destruction forestière, de limites de pêche, etc. Quel est

Les nombreuses atteintes à la biodiversité et à l'environnement pourraient à terme provoquer la destruction de l'humanité. Ainsi, la France doit mettre en oeuvre toutes les politiques environnementales nécessaires pour limiter l'impact des activités humaines à un niveau permettant à l'humanité de disposer des fonctions essentielles de la biosphère.

La dégradation de l'environnement, le changement climatique et le développement non durable comptent parmi les menaces les plus imminentes et les plus graves qui pèsent sur le droit à la vie des générations actuelles et futures. Nous souhaitons ainsi rappeler l'impact de nos décisions actuelles et leurs conséquences sur les capacités des générations futures à vivre dans de bonnes conditions environnementales. Ce droit à un environnement sain, dans lequel on peut inclure le droit à l'eau, à un air non pollué, aux bénéfices de la biodiversité, a été reconnu en France et est inscrit dans la Charte de l'environnement de 2004. Il convient cependant d'en renforcer la portée juridique en l'érigeant en principe constitutionnel inscrit à l'article 1 de la Constitution.

du préambule de la Charte de l'environnement de 2004, qui dispose que, « afin d'assurer un développement durable, les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures et des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins ». Les choses sont claires, l'avis est donc défavorable.

Le principe de non-régression protège les droits des générations futures en renforçant les exigences écologiques dans la prise de décision. L'effectivité d'un droit humain à l'environnement ne devient réalité l'établissement d'une garantie juridique assurant que chaque avancée pour la préservation de l'environnement ne peut être remise en cause. Ce principe n'implique pas une impossibilité d'action de la part des autorités, mais crée une obligation positive, notamment pour le législateur, de ne pas dégrader les avancées écologiques. En dépit de l'urgence climatique, certaines décisions législatives ou réglementaires effet moins-disantes au niveau environnemental ; ce retour sur la protection de l'environnement et de la biodiversité nous semble insupportable. Au vu des dernières décisions qui ont permis, par exemple, au juge de valider un retour en arrière sur la limitation des néonicotinoïdes, il est essentiel d'inscrire dans la Constitution que, à défaut de faire plus, on ne peut plus se permettre de faire moins.

La proposition du Président de la République d'inscrire à l'article 1 de la Constitution l'engagement du pays en faveur de l'environnement et dans la lutte contre le dérèglement climatique nécessite, pour avoir quelque chance de succès, d'associer à cette démarche vertueuse l'ensemble de nos concitoyens et de nos institutions. Les Françaises et les Français se sont largement exprimés sur ce sujet, notamment lors du grand débat ou par l'intermédiaire de la Convention citoyenne pour le climat, souhaitant recourir à un référendum.

des espaces naturels contribuant aux objectifs de maintien de la diversité biologique, porteurs de services écosystémiques rendus par la nature. Il existe donc un lien intime et subtil qui relie environnement et territoires,

Dans cette approche environnementale nous devons mettre toutes les chances de notre côté et corriger le modèle de société qui est le nôtre en nous souvenant de ce que disait Hubert Reeves : « Actuellement, l'homme mène une guerre contre la nature. S'il gagne, il est perdu. » Quel

Je suis persuadé que cet amendement va faire l'unanimité sur ces travées ! Le groupe Écologiste-Solidarité et Territoires appelle à une transformation majeure du processus législatif en adoptant, pour l'ensemble des textes de loi sur l'environnement, l'obligation de la publication d'une étude d'impact climatique avant leur examen parlementaire. La France ne dispose pas de moyens permettant de piloter et de mesurer l'impact des lois au regard de l'objectif carbone fixé pour 2050. Il est donc indispensable d'intégrer une évaluation des impacts climatiques dans le processus de conception des politiques publiques. Le Haut Conseil pour le climat, dans un rapport publié le 18 décembre 2019, recommandait de mettre en place une telle évaluation climatique des projets et propositions de loi.

qui placerait la France en cohérence avec ses ambitions de protection de l'environnement et de lutte contre le réchauffement climatique.

d'une étude d'impact, quelle que soit la nature de celle-ci. Cela devrait suffire à satisfaire votre intérêt pour cette question. Avis défavorable.

Cette autorité constitutionnelle indépendante veillerait au respect par l'État et par ses administrations, ainsi que par l'ensemble des personnes morales, de cet engagement écologique essentiel. Le contenu de la loi organique s'y rapportant, comprenant notamment la procédure de nomination, se calquerait sur celui qui s'attache au Défenseur des droits. Nous avons pu observer combien, ces dernières années, le travail du Défenseur des droits a permis d'alerter les responsables sur un certain nombre de conséquences et d'éviter des violations des droits des citoyens. Considérant qu'un principe constitutionnel n'a de sens que s'il bénéficie aux citoyens, nous souhaiterions voir l'émergence de ce Défenseur.

Par ailleurs, il pourrait être utile, en particulier, de créer un dispositif de médiation chargé de régler à l'amiable les litiges qui peuvent naître entre l'administration et les citoyens en matière de protection de l'environnement. En effet, le droit de l'environnement est extrêmement complexe et il est toujours

appelée à se prononcer, par exemple, sur les projets de loi relatifs à l'environnement. Je rappelle qu'il existe un Conseil économique, social et environnemental dont c'est le rôle et que nous venons de réformer. Enfin, je note que la Enfin, je note que la protection du droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, consacré par notre Charte de l'environnement, entre dans les missions du Défenseur des droits,

À cet égard, l'utilisation du terme « biodiversité » a le mérite de faire preuve de clarté, au contraire de celui de « diversité biologique ». La biodiversité est définie par la Convention sur la diversité biologique comme « la variabilité des êtres vivants de toute origine y compris, entre autres, les écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partie

géographique. On ne peut donc accepter que nos parcs naturels soient dénaturés par l'installation de structures, comme les éoliennes ou des antennes relais, qui peuvent parfois menacer la biodiversité en artificialisant les milieux naturels.

Par ailleurs, il serait étrange d'inscrire dans l'intitulé le terme « biodiversité », alors que nous venons de préférer inscrire à l'article unique la mention « diversité biologique » pour être en parfaite cohérence avec la Charte de l'environnement. Enfin, s'agissant de la référence au paysage naturel, la commission des lois craint une confusion. Le droit constitutionnel de l'environnement est aujourd'hui centré d'abord sur la protection de la santé de

produit de siècles d'histoire et, en particulier, de la diversité des pratiques agricoles et sylvicoles. Pour ces raisons, la commission des lois a souhaité vous demander de retirer votre amendement ; à défaut, son avis serait défavorable. Je

Sûrement à l'exécutif, monsieur le garde des sceaux, qui, avec un cynisme assumé, n'a pas pris les voies et moyens pour parvenir à un vote conforme entre les deux chambres en dramatisant la situation politique par le recours, officiellement, au référendum à six mois de l'échéance présidentielle, tout en espérant, officieusement, que celui-ci ne puisse avoir lieu. Monsieur le garde des sceaux, la manipulation de l'opinion et l'instrumentalisation du Parlement ne sont pas à votre honneur

pour s'opposer institutionnellement à cette tentative de modification de l'article 1, tout en décrédibilisant un processus participatif qui méritait manifestement plus de reconnaissance de votre part. Devant cette Devant cette situation provoquée par la majorité présidentielle et par la droite sénatoriale, nous vous laisserons dos à dos, ... en nous opposant au texte issu des débats de ce soir, qui se conclut par un crash politique incompréhensible pour nos concitoyens. La protection de la planète, la notion de biens communs, défendue par notre collègue Nicole Bonnefoy, méritaient sûrement mieux, dans l'esprit des accords de la COP21 que nous avons porté durant le quinquennat précédent. La parole pour explication de vote. Dans certains cas, notre Haute Assemblée bénéficie d'une forme de dernier mot. Comme les lois relatives au Sénat, la Constitution ne peut être modifiée sans l'aval des sénatrices et sénateurs. Ce soir, nous faisons le constat d'un désaccord entre les deux chambres sur le contenu du texte à soumettre aux Françaises et aux Français par la voie référendaire.

Nous passerons donc, cette réécriture, d'une prétendue incertitude quant aux effets de la révision initialement proposée à une apparente certitude sur l'absence de portée juridique de la rédaction qui sortira du Sénat.

soutenir le « oui » au projet de révision dans la rédaction que nous votons ce soir consisterait à convaincre les citoyens de se rendre aux urnes pour approuver une révision constitutionnelle dont l'auteur affirme qu'elle n'aurait pas de portée. Nous le comprenons mal, au regard de l'objectif, partagé, de mobiliser autour d'un référendum les citoyens français sur l'enjeu en question. Pour ces raisons, le groupe RDPI votera majoritairement contre la version proposée par la majorité sénatoriale, laquelle ne nous paraît pas suffisamment protectrice au regard de notre ambition. Quant

fruit d'une proposition de la Convention citoyenne sur le climat. Je ne reviendrai pas sur les circonstances ayant conduit à cette proposition de révision. Je tiens simplement à rappeler que, à l'heure où la légitimité de nos institutions est parfois contestée, recourir au tirage au sort apparaît comme une bien mauvaise idée. Reprendre, sans filtre, une proposition est un affaiblissement des pouvoirs du Constituant. Votre inflexibilité quant au texte soumis à l'examen du Parlement, monsieur le garde des sceaux, confirme cet affaiblissement et nous le déplorons solennellement. Nous voyons d'ailleurs bien dans quel piège le Gouvernement s'est placé : vous soumettez à la discussion de la représentation nationale un texte qui n'a pas vocation à évoluer. Quelle conception du débat parlementaire vous faites-vous donc ? Les propos rapportés de l'Élysée le démontrent : il n'y aura pas de référendum, parce que cette révision n'était qu'un moyen facile de donner des gages aux conventionnels, tout en se défaussant sur le dos du Sénat. La manipulation est grossière et aventureuse. Qu'a voulu faire notre groupe sur ce texte ? La droite républicaine a défendu ce soir une écologie de progrès au service de tous nos concitoyens. Cette vision de l'écologie ne peut être que conciliée avec d'autres déterminants de notre prospérité, notamment le développement économique et le progrès social. C'est, du reste, ce que rappelle l'article 6 de la Charte de l'environnement dans la définition qu'il donne du développement durable. C'est cette conciliation que notre groupe a voulu assurer dans la révision constitutionnelle qui nous était soumise, et je tiens tout particulièrement à saluer le travail de nos deux rapporteurs François-Noël Buffet et Guillaume Chevrollier. La modification de l'article 1 adoptée par notre assemblée lève ainsi toute ambiguïté juridique, car nous ne voulons pas, comme le rapporteur l'a soutenu, constitutionnaliser le doute. Elle permet aussi de renvoyer expressément à la Charte de l'environnement. Le travail du Sénat est ainsi bénéfique à double titre : d'une part, nous introduisons à l'article 1 de notre norme suprême la question environnementale tout en évitant, d'autre part, de laisser au juge constitutionnel un trop fort pouvoir d'interprétation au détriment de l'action des entreprises et des collectivités. La balle est désormais dans le camp du Gouvernement et de sa majorité. À vous de prouver que toute cette opération n'était pas seulement un jeu cynique visant à contester les droits souverains du Parlement. Bien entendu, nous voterons le texte ainsi modifié par le Sénat.

Nous voterons contre une proposition qui ne prend pas la mesure de l'urgence climatique. Nous voterons contre un positionnement caricatural face à la priorité de l'urgence écologique. En revanche, nous aurions souhaité voter pour garantir la préservation de l'environnement et de la diversité biologique, la lutte contre le dérèglement climatique.

Toutefois, mes chers collègues, vous qui êtes si attachés au respect de la démocratie représentative et de la consultation citoyenne, vous devriez tout au moins

est une forme de bien-pensance que nous ne pouvons pas accepter

demande plus la parole ? ... Je mets aux voix, modifié, l'ensemble du projet de loi constitutionnelle. En application de l'article 59 du règlement, le scrutin public ordinaire est de droit. Il va y être procédé dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert.